Sur le fond, c'est une problématique bien plus large que nous abordons. La question est simple : allons-nous continuer longtemps à appliquer ce modèle du tout-plastique, du tout-jetable et de l'exploitation des ressources naturelles jusqu'à plus soif, pour garantir les profits de quelques grands groupes industriels ? Allons-nous continuer d'avancer, tête baissée, vers la sixième extinction de masse des espèces et de supporter qu'il y ait dans nos océans plus de plastique que de poisson ? Et pourquoi tout cela ? Pour conforter un système libéral fondé sur l'exploitation des hommes, sur la surproduction, donc sur la surconsommation, antinomique avec la préservation de l'humanité et l'intérêt des peuples. Le groupe CRCE propose une démarche cohérente. D'abord, nous assumons notre conviction : il est urgent de sortir de ce modèle cannibale, comme le nommait un ancien ministre de l'environnement. Pour cela, nous pointons un horizon : en 2040, nous devrons être sortis du modèle du plastique, donc du pétrole. Cet engagement est cohérent avec la date butoir de 2040 posée pour l'exploitation des énergies fossiles. Il nous semble ainsi cohérent de poser, à cette date, l'interdiction du plastique unique, qui engendre une utilisation de pétrole particulièrement inutile 3,2 grammes de pétrole dans un gobelet, 10 centilitres de pétrole dans une bouteille d'un litre. Il s'agit d'envoyer un signal clair, à la fois à la population et aux industriels, dans une temporalité supportable qui permettra d'accompagner les secteurs concernés. En effet, si cette transition est bien menée, elle promet un gisement d'emplois non délocalisables. Il faut tenir sur nos deux jambes : un discours ferme de changement, mais aussi un accompagnement des territoires et des secteurs appelés à se transformer pour ne pas créer demain de nouvelles friches industrielles, avec le lot de vies brisées que nous avons déjà connu. Les interdictions plus ponctuelles que nous proposons sont autant de cailloux semés pour signifier que les temps changent, que l'opinion publique évolue et qu'il convient d'acter ce changement de paradigme, quitte à rediscuter de ces échéances en cours de route. C'est la démarche que nous avons engagée sur le glyphosate, les OGM et autres pesticides ou perturbateurs endocriniens. Il convient en tout état de cause de poser des actes politiques forts ; nous espérons donc que nos amendements seront adoptés. La Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, que diront ceux qui après nous viendront ? Que nous n'avons rien fait, alors que nous savions. Le plastique est problématique. C'est le matériau à la durée d'usage la plus courte et à la durée de vie la plus longue. Le plastique ne se décompose pas ; il se fractionne, mais reste toujours du plastique. La France produit actuellement 5 millions de tonnes de plastique par an ; cette production est en augmentation. Or 75 % du plastique produit devient un déchet dans un délai extrêmement court.

: il n'y a pas d'autre solution ! Les signaux s'accumulent, notamment quant aux risques pour la santé ; les preuves scientifiques sont là. Si l'on attend encore pour agir, il sera trop tard ! Les connaissances s'empilent à grande vitesse et elles disent toutes la même chose

Qu'allons-nous laisser dans la nature après nous ? Des marques de notre civilisation, le bitume et le plastique, certainement. Nous ne pouvons plus sacrifier l'écologie dans les actes. Je vous propose d'avoir de l'audace et d'inscrire dans ce texte notre volonté de rompre avec des pratiques qui sont des non-sens écologiques. Avec tout ce que nous savons, comment continuer de permettre qu'on enveloppe entièrement de plastique un concombre bio ? bio ? En tant que législateur, notre vision n'est pas purement économique ; elle doit exprimer l'intérêt général. Il nous faut montrer que l'ère de l'utilisation irraisonnée du plastique est révolue et que ce sont des pratiques d'un autre âge.

Beaucoup d'amendements ont été déposés par divers collègues sur la question de l'extension ou du report des interdictions figurant déjà dans notre droit en ce qui concerne la mise à disposition ou la distribution d'objets en plastique à usage unique.

L'approche de la commission a été double. D'une part, elle n'a pas souhaité étendre des interdictions qui constitueraient des surtranspositions du droit européen et dont les impacts n'auraient pas été évalués.

Au contraire, la commission a fait le choix de lutter de manière globale contre les suremballages, via la mise en place par les pouvoirs publics d'une trajectoire pluriannuelle de réduction de la mise sur le marché d'emballages, l'obligation pour les entreprises qui suremballent de réaliser des plans d'éco-conception et de prévention, et l'instauration d'un malus financier sur le suremballage.

des déchets : 100 % de plastique recyclé en 2025, une réduction de 50 % de la mise sur le marché d'emballages à usage unique d'ici à 2030, puis à nouveau de 50 % entre 2030

aujourd'hui les sacs en plastique de faible épaisseur, mais elle autorise toujours les sacs en plastique épais, sous prétexte qu'ils sont réutilisables. Je viens de Nouvelle-Calédonie : l'endroit du monde qui compte la plus grande biodiversité, après Madagascar ; un territoire exceptionnel. Mais la Calédonie n'échappe pas à la pollution des sacs plastiques, des canettes et des bouteilles en plastique. La mangrove en est recouverte, tout comme les bords des routes et les rivières. Partout du plastique, du plastique, du plastique Comme nous avons la compétence sur l'environnement, nous avons enfin interdit les sacs en plastique dans les commerces

Labbé, pour présenter l'amendement n° 674 rectifié . Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape en interdisant l'ensemble des sacs plastiques utilisés dans les points de vente. Ces sacs font partie des déchets que l'on retrouve en

Nous avons tous en tête les tristes images de milieux marins envahis par des sacs plastiques. La loi de transition énergétique a interdit la mise à disposition en caisse des sacs en plastique dits « à usage unique

Eh bien, dans les magasins, cela fonctionne ! Les consommateurs jouent le jeu, par choix ou par obligation, mais c'est bien notre rôle que de mettre en place de telles obligations. Si cette mesure a permis de réduire la consommation de sacs en plastique, les sacs épais sont encore distribués massivement et ne sont que trop peu réutilisés. Ces sacs vident en partie de sa substance l'interdiction prévue et limitent donc fortement fortement son efficacité. De plus, les dispositifs de compostage domestique étant encore trop peu développés, de même que la collecte des déchets organiques auprès des particuliers, les sacs hors caisse compostables sont souvent jetés dans les ordures ménagères. Ils peuvent également perturber les filières de tri et de recyclage. En outre, la mention « biodégradable » sur ces sacs peut induire en erreur le consommateur, qui peut penser que ce sac se dégrade naturellement lorsqu'il est jeté dans l'environnement, alors qu'il ne se décompose en réalité que dans des conditions précises. Des alternatives, comme le papier, paraissent bien plus écologiques et facilement substituables. Cet amendement vise donc à interdire la mise à disposition de l'ensemble des sacs plastiques. La date d'entrée en vigueur de cette interdiction, prévue en 2022, doit permettre aux entreprises de s'adapter.

M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous proposons de traduire la directive européenne récente sur le plastique et de corriger le code de l'environnement en conséquence. En effet, la directive européenne ne prévoit pas, comme en droit national, d'exception à la mise sur le marché de produits en plastique à usage unique pour les plastiques compostables ou biosourcés. La directive européenne 2019/904 est particulièrement claire à ce sujet. En effet, pour justifier de sa définition du plastique, il est indiqué : « Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d'origine biologique, fossiles ou synthétiques n'existent pas naturellement dans l'environnement et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s'appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d'origine biologique et biodégradables, qu'ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. une interdiction pure et simple que nous soutenons. En effet, les associations nous ont alertés sur le fait que, à ce jour, aucun produit fini n'a encore été approuvé comme biodégradable dans l'environnement marin. En outre, la norme européenne de compostage des emballages garantit seulement la biodégradation des emballages dans des conditions industrielles, et non domestiques. Par ailleurs, remplacer le plastique conventionnel par du bioplastique impliquerait l'utilisation de centaines d'hectares de terres pour sa production, ce qui aurait pour conséquences l'appauvrissement des terres, la création de conflits de terre, une possible perte d'habitats naturels et l'utilisation de ressources importantes en eau, ce qui ne nous semble évidemment pas souhaitable. Ces exceptions dans le code de l'environnement sur les interdictions de mise sur le marché de produits en plastique à usage unique ne sont donc ni justifiées ni pertinentes ; leur maintien placerait la France en contradiction avec le droit européen.

C'est une lutte dans laquelle la France, deuxième puissance maritime mondiale, doit être en pointe. Lors du sommet du G7, à Biarritz, le Président de la République s'est vu remettre, au nom du département des Pyrénées-Atlantiques, par notre collègue Max Brisson, accompagné du maire de Biarritz et du président de la région Nouvelle-Aquitaine, un mémorandum sur l'avenir des océans élaboré par les collectivités dans le

Aussi, M. Brisson propose d'étendre la fin de la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, des sacs plastiques à usage unique aux sacs biodégradables et biosourcés, qui ont un impact majeur sur l'environnement marin. Je partage son opinion.

amendement vise donc à mettre en cohérence les dispositions françaises avec le droit européen récemment modifié en matière de mise à disposition et d'usage de certains produits en plastique.

Mme Jacky Deromedi. Les déchets en plastique ont un impact considérable sur l'environnement et, en particulier, sur les océans. La Commission européenne avait conclu, dans son plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire, que le problème de l'augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de ces déchets dans l'environnement devait être résolu afin d'instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement entend répondre à cet objectif. Aux termes de son article premier, cette directive « vise à prévenir et à réduire l'incidence l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu'à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur Parmi les mesures contenues dans cette directive figurent la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et l'interdiction de certains autres. Les États membres ont jusqu'au 3 juillet 2021 pour adopter les mesures nécessaires. Afin de respecter la directive européenne, le présent amendement vise à fixer au 3 juillet 2021 l'interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables, ainsi que des pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique.

Cet amendement vise à mettre fin à l'usage du polystyrène expansé pour les emballages alimentaires. Le polystyrène expansé est souvent utilisé pour emballer des produits de restauration à emporter. Les conditions de son usage, généralement nomade et à l'extérieur, sont telles que ces emballages sont trop souvent jetés directement dans l'environnement et, en tous les cas, très peu triés et recyclés. Ils ont donc un impact direct sur l'environnement et sont source de pollution, notamment pour les milieux marins. Il est donc essentiel de prévoir une interdiction, d'autant plus que ces contenants peuvent être facilement remplacés par des alternatives réutilisables et éco-conçues. La date d'entrée en vigueur proposée de cette mesure, à savoir le 1 janvier 2021, permettra aux entreprises de s'adapter. Cette interdiction est conforme à la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. En effet, cette directive dispose que, « compte tenu de la prévalence élevée des déchets sauvages en polystyrène expansé dans le milieu marin et de la disponibilité de produits alternatifs, il y a lieu de limiter également les récipients pour aliments, les récipients pour boissons et les gobelets pour boissons à usage unique en polystyrène expansé

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.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

tel que fixé dans la directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

Alors que l'article 10 prétend traduire en droit les obligations liées à la directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, certains oublis nous semblent regrettables. En effet, cet article se concentre sur le plastique oxodégradable, alors que les avancées de la directive sont bien plus importantes.

nous considérons qu'il convient d'aller vers une interdiction pure et simple de l'ensemble des emballages et des contenants en polystyrène expansé, une interdiction encouragée par le droit européen, qui permettrait de mettre fin à ce fléau des emballages non recyclables, pour lesquels une alternative existe. Il faut que le Parlement pose des actes forts pour la protection de notre écosystème et des océans. Nous ne pouvons plus tolérer cette pollution aux conséquences dramatiques. En tout état de cause, ce projet de loi sur l'économie circulaire ne peut fixer des ambitions en deçà du droit européen.

en plastique dans un champ très large de lieux publics. Or cette disposition paraît sans bien-fondé sanitaire ou environnemental. L'eau est un produit de première nécessité : près de 95 % des Français achètent de l'eau en bouteille. L'eau en bouteille est uniquement destinée à être bue, alors que l'eau du robinet est destinée à 99 % à des usages ménagers. L'article 10 pénalise donc tous les Français qui la consomment, sans apporter de réponse crédible et rationnelle aux objectifs de ce projet de loi. Au demeurant, Au demeurant, précisons que, dans sa rédaction issue des travaux des commissaires, l'article 10 fragiliserait un tissu économique de 12 000 emplois « non délocalisables » situés majoritairement en zone rurale ou en zone de montagne.

Adoptée sans étude d'impact préalable, cette mesure arbitraire aurait pour effet un moindre accès du public à l'eau minérale naturelle, sans traiter de la question des autres boissons sucrées ou alcoolisées, qui peuvent être délivrées de la même façon ou à titre onéreux et qui présentent pourtant un bilan sanitaire bien moins favorable. Cette mesure ne permet pas non plus d'appréhender l'ensemble des situations de distribution gratuite de bouteilles d'eau plate en plastique qui ne sont pas compatibles avec la mise à disposition d'eau du robinet. Enfin, cette disposition risque de pénaliser le public, qui, partout où il se voit actuellement proposer des bouteilles d'eau plate en plastique, se verra demain proposer des bouteilles d'eau minérale payante. Au contraire, il convient d'encourager la consommation d'eau sous toutes ses formes et de la rendre accessible par le plus grand nombre.

Il n'y a donc pas de raison de mettre à disposition des bouteilles individuelles, dont le bilan écologique est catastrophique. Trois gorgées d'eau et combien de temps pour que la bouteille se dégrade ? Entre 100 et 1 000 ans Dans le Pacifique, la faune meurt du plastique : il s'en retrouve dans tous les organismes vivants. Il existe même un continent entier dans cet océan, grand comme six fois la France, constitué uniquement de matières plastiques.

Il n'y a d'ailleurs pas plus de raison d'autoriser les bouteilles gratuites que les bouteilles payantes : l'impact écologique est le même. Quand on a interdit la cigarette dans les lieux publics, a-t-on fait la distinction entre les cigarettes avec filtre

Son application fragiliserait les territoires ; les mairies et les associations culturelles, sportives ou caritatives se trouveraient en effet privées d'un soutien indispensable sans réelle solution de remplacement pour leurs événements. La plupart des situations de distribution gratuite ne permettent pas l'utilisation d'un autre contenant. De plus, la substitution par l'eau du robinet n'est généralement pas possible pour des raisons logistiques- absence de fontaines, nécessité de gobelets ... -ou hygiéniques. Durant les épisodes caniculaires, cet été, nombre d'établissements ont mis des bouteilles d'eau à la disposition de leurs clients ou du public, notamment dans les métros et les trains. La distribution aux participants de festivals, salons, manifestations culturelles,

parole est à Mme Nicole Duranton. L'information selon laquelle la distribution gratuite d'eau potable du robinet est obligatoire pour les établissements de restauration est bien connue de l'ensemble des citoyens, qui usent de cette disposition Il ne paraît donc pas utile de contraindre par la loi les établissements à réimprimer leur carte, ce qui représenterait par ailleurs un coût économique et écologique certain, ou à afficher cette information déjà connue de tous.

qui interdit, à compter du 1 janvier 2020, la distribution gratuite de bouteilles d'eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, et qui rend obligatoire pour les restaurants la mise à disposition

Merci, monsieur le président

? Le véritable cercle vertueux et circulaire de l'eau doit être la protection de la ressource. C'est la raison pour laquelle nous luttons farouchement contre les pesticides

Cet amendement vise à interdire les bouteilles en plastique pour la consommation d'eau et de boisson dans les administrations via la commande publique. Comme cela a été dit à plusieurs reprises au cours des débats, nous pensons que l'État et l'administration doivent être exemplaires en matière de réduction des déchets et, de manière plus générale, de développement d'une économie circulaire efficace.

Le 20 septembre dernier, la justice européenne a confirmé la classification du bisphénol A comme perturbateur endocrinien, classification qui avait été décidée en juillet 2017 par l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA,

tout perturbateur endocrinien dans les plastiques qui sont actuellement au contact des populations. On le sait, ces substances chimiques sont extrêmement toxiques et nocives pour la santé des êtres humains,

Merci, monsieur le président d'emballages. Certaines régions du monde ont adopté ces derniers mois des restrictions similaires à celle que tend à prévoir le présent amendement : la ville de Berkeley aux États-Unis a voté l'obligation d'utiliser des articles de cuisine réutilisables pour la restauration sur place à partir de juillet 2020 ; les îles Baléares en Espagne ont prévu l'interdiction des récipients à usage unique pour les repas pris sur place

la restauration rapide produit chaque année 180 000 tonnes d'emballages et ne trie que très rarement ses déchets, au mépris de la réglementation en vigueur. Lorsqu'un repas est pris sur place, les emballages pourraient aisément être remplacés par des contenants réutilisables. Il vous est donc proposé d'interdire l'utilisation d'emballages jetables pour les repas pris sur place, afin de mettre fin à des pratiques qui sont désormais dépassées.

Nous visons plus particulièrement les établissements de restauration rapide, qui produisent chaque année 183 000 tonnes d'emballages. Le délai de cinq ans envisagé pour y parvenir nous semble largement suffisant pour permettre à ces établissements d'anticiper et de s'adapter à cette nécessaire

Le scrutin est ouvert.

Actuellement, plus de 150 millions de tonnes de plastique sont déjà présentes en milieu marin. Si les États et les citoyens n'agissent pas, les océans pourraient contenir une tonne de plastiques pour trois tonnes de poissons d'ici à 2025. Ces chiffres, nous ne les inventons pas. Ils figurent tout simplement sur le site du ministère de l'environnement. Nous considérons donc que nous devons aller beaucoup plus loin dans les interdictions et limiter tous les produits plastiques à usage unique, qui sont un non-sens environnemental. Aujourd'hui, c'est la stratégie des petits pas. En tout, une dizaine de catégories de produits est concernée. Parmi elles, les pailles, les touillettes, les couverts, ou encore les gobelets et les cotons-tiges.

date est cohérente, puisqu'il s'agit de l'échéance que nous nous sommes fixée pour sortir de l'exploitation des hydrocarbures et donc du pétrole. L'interdiction à cette date de plastique à usage unique semble donc à la fois crédible et cohérente. Le délai est largement suffisant pour que les industriels puissent s'adapter à ce choix de société. Ces industriels, mais également les territoires, doivent être accompagnés dans ces mutations technologiques par les pouvoirs publics, et il convient que la transition écologique soit réellement le gisement d'emploi que nous attendons tous, y compris les salariés de ces usines. Déjà aujourd'hui, des alternatives existent : de l'inox ou du bois pour les couverts, des récipients en verre pour les aliments, des mugs en terre cuite pour les boissons, des gourdes en lieu et place des bouteilles en plastique. Nous pourrions d'ailleurs utiliser largement ces dernières au Sénat. une gourde à chaque sénateur en début de mandat pour éviter l'usage des bouteilles et des verres en plastique ? Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la volonté politique pour favoriser ces filières innovantes en plaçant un véritable objectif compréhensible, en accompagnant les entreprises, mais en fixant un cap clair, fin de l'exploitation des énergies fossiles et donc à celle du plastique à usage unique. Quel Nous partageons bien sûr vos objectifs. En réalité, cher collègue, votre amendement est quasiment satisfait par les objectifs ambitieux que nous avons adoptés au début du texte. Je les rappelle : 100 % des plastiques recyclés en 2025, une réduction de 50 % des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché en 2030, et encore de 50 % en 2040 par rapport à 2030. L'avis de la commission est donc défavorable.

la mise sur le marché d'emballages à usage unique en plastique. Nous estimons que ce que vous demandez à travers cet amendement est quasiment satisfait.

de microplastiques dans différentes catégories de produits de consommation courante ou à usage professionnel, étendant ainsi l'interdiction déjà en vigueur des microplastiques dans les cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage adoptée dans la loi Biodiversité. Il se situe dans la lignée des recommandations de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, qui préconise de mettre fin progressivement à l'ajout de microplastiques dans un certain nombre de produits, comme les cosmétiques, les peintures, les détergents, mais aussi les fertilisants agricoles. Selon cette agence, dans l'Union européenne, la quantité de microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits qui s'infiltrent dans l'environnement chaque année est estimée à environ 36 000 tonnes par anCes microplastiques sont ainsi une source majeure de pollution des milieux, notamment des milieux aquatiques. S'il reste encore des incertitudes quant à leur impact sur la santé, on peut largement présupposer que ces particules, qui se retrouvent dans des produits alimentaires

ne cessent d'ailleurs de s'accroître, sans qu'elle dispose des moyens de les assurer. Il faut donc profiter de ce texte pour agir rapidement sur le sujet. Un décret pourra préciser les catégories de biens concernés et la date d'entrée en vigueur de l'interdiction pour chaque catégorie, catégorie, afin de s'adapter à chaque filière en fonction de sa possibilité de développer rapidement des alternatives, en vue de rendre applicable cette interdiction pour les entreprises. l'avis de la commission ? Nous comprenons parfaitement votre demande, cher collègue, et nous la partageons. La difficulté tient à la manière dont l'amendement est présenté : une telle interdiction ne peut être prononcée ainsi. Le champ de cette interdiction est potentiellement très et pourrait concerner un grand champ de produits de consommation courante, mais aussi à usage professionnel. L'impact a-t-il été mesuré ? L'effet serait en outre immédiat. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Cet amendement vise à interdire la mise sur le marché de bouteilles en plastique de moins de 75 centilitres. Il s'agit de mettre un terme à ce type de contenant à usage unique, qui semble en totale contradiction avec la préservation de l'environnement. Nous devons changer nos habitudes face à la dérive qui est la nôtre d'utilisation de bouteilles d'eau de petit format. C'est une gabegie, considérant que leur usage, très éphémère, n'est parfois que de quelques minutes. C'est aussi mettre fin à une certaine forme d'addiction à la facilité. Certains de nos concitoyens ont déjà adopté d'autres contenants, comme des gourdes, mais ce n'est pas suffisant. Le maître mot pour lutter contre la pollution plastique et pour lutter contre ce gaspillage, c'est la réduction à la source, ce qui me paraît évident. Or quel exemple plus éloquent qu'une bouteille en plastique de 25 centilitres, par exemple, tellement vite bue, tellement vite jetée ? Il faut amorcer le basculement de notre société du jetable vers une société plus respectueuse de nous-mêmes, tout simplement. Nous n'avons plus le temps d'attendre que tout le monde en soit persuadé, au détriment de l'environnement et de notre santé.

M. Éric Gold. Nous avons déjà souligné l'importance de limiter les déchets en amont, par exemple en limitant la production de plastique. Nous vous proposons donc d'interdire une forme de gaspillage qui participe chaque jour à accroître notre production de déchets. En effet, 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour en France. cette consommation se justifie, des efforts peuvent être faits pour la limiter drastiquement. C'est le cas notamment des toutes petites bouteilles en plastique qui se multiplient, contre toute logique et à rebours de la prise de conscience de nos sociétés. Les bouteilles de 20 centilitres contiennent 20 grammes de plastique, soit un gramme Cet amendement s'inscrit donc dans un souci d'effort commun pour limiter notre impact sur l'environnement, à la fois en termes d'utilisation de matières premières et de production de déchets. Quel

Je partage totalement votre ambition de lutter drastiquement contre la pollution plastique. J'ai proposé plusieurs solutions, et ce projet de loi en contient beaucoup. Un jour, je suis convaincue que nous pourrons et devrons nous passer totalement des bouteilles en plastique.

Vous avez raison, nous devons nous y préparer, préparer notre industrie à une telle transformation et anticiper les conséquences très lourdes que cela pourrait avoir sur la façon de transporter, d'emballer et de consommer les boissons. Une telle décision doit être nourrie par une réflexion approfondie que nous devons lancer dans la perspective du débat à l'Assemblée nationale.

Le scrutin est ouvert.

En France, des initiatives intéressantes peuvent être soulignées. Ainsi, depuis le 1 janvier 2017, plus aucun magasin Biocoop ne distribue d'eau en bouteilles plastiques. Nous pensons donc qu'il convient aujourd'hui, pour l'exemplarité de notre pays, de franchir un cap supplémentaire, afin de lutter efficacement contre la pollution liée au plastique.

doit rester la réduction à la source des déchets, et donc le développement des alternatives au plastique à usage unique et aux autres matériaux non réutilisables. Il s'agit également de donner un coup de pouce à la mise en place En effet, l'établissement d'un quota d'emballages réutilisables permettra non seulement de préserver les gammes d'emballages réutilisables d'ores et déjà mises en oeuvre, mais également de s'appuyer sur les infrastructures existantes pour développer de nouveaux circuits de réutilisation des emballages à destination des consommateurs. Cette mesure est « euro-compatible », puisque la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages donne la possibilité aux États membres de définir « des objectifs qualitatifs et quantitatifs » et « un pourcentage minimal d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages nous inscrivons donc clairement ici dans le cadre d'une transposition effective de la directive européenne. Nous proposons que ces quotas soient établis par décret, après consultation des parties prenantes. Fixer à 2021 l'échéance pour l'établissement des premiers quotas permet, en outre, de laisser le temps au secteur de s'adapter.

Les marges de progression en France sont donc importantes, et la transition vers un mode de conditionnement et de distribution des boissons plus durable peut se faire dans les prochaines années, à condition que les signaux politiques et économiques adressés soient les bons. Il est à cet égard nécessaire d'intégrer dans la loi des mesures susceptibles de garantir un déploiement progressif des solutions de réemploi et de réutilisation des emballages. Cet amendement vise à fixer un objectif minimal de pourcentage d'emballages réutilisables mis sur le marché à partir de 2022. Cette mesure est permise par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui donne la possibilité aux États membres de définir « des objectifs qualitatifs et quantitatifs » et « un pourcentage minimal d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages ». Quel

Dans la pratique, sa mise en oeuvre imposerait une certaine conception des emballages pour qu'ils soient réutilisables, ce que proscrit la directive. Il me semble utile de souligner que les autorités danoises ont mis en oeuvre, il y a plusieurs décennies, un dispositif comparable à celui de ces amendements.

L'État a pris l'engagement de tendre vers 100 % de plastique recyclé et l'Union européenne vise l'incorporation de 10 millions de tonnes de matières plastiques recyclées à l'horizon 2025. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'actualiser notre arsenal juridique. Le présent amendement crée ainsi une obligation d'incorporation progressive de matières premières recyclées par segment d'activité

Cette mesure aurait une incidence beaucoup plus importante sur l'environnement que le simple déploiement d'une consigne pour recyclage, en permettant de privilégier la prévention la production de déchets ou le réemploi.

défavorable. J'insiste encore une fois sur l'importance de savoir de quoi on parle et d'établir des études d'impact rigoureuses pour nourrir les décisions des responsables politiques que nous sommes.

Les débris des ballons qui éclatent retombent sur terre et en mer. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, les débris de ballons sont dans le « top 10 » des déchets récréatifs retrouvés sur le littoral. Leurs fragments sont également retrouvés dans les estomacs d'animaux marins. En France, ce sont près d'un million de ballons qui s'envolent chaque année. Ils peuvent monter jusqu'à huit kilomètres d'altitude et leurs débris se retrouvent dans des périmètres très larges. Cet amendement vise à limiter la pollution liée à l'éclatement des ballons

C'est pour enrayer cette pollution que des villes comme Brighton, en Grande-Bretagne, ou Victoria, en Australie, ont interdit les lâchers de ballons. Depuis juillet dernier, un arrêté préfectoral les interdit également dans le département de Saône-et-Loire.

vise ici les microplastiques qui constituent une composante, un ingrédient du produit, à la différence des microplastiques qui sont créés au cours du cycle de vie d'un produit en raison de l'usure ou d'un déversement accidentel

et ne dépasse pas 5 millimètres. Elles sont composées de polyéthylène, mais aussi de polypropylène, de polytéréphtalate d'éthylène, de polyméthylméthacrylate ou de nylon. Les microbilles ne sont pas uniquement utilisées pour leurs vertus exfoliantes et nettoyantes, mais également pour en tant qu'agent de polissage,

pour être retenues par les filtres des stations d'épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d'eau, pour finir leur course dans l'océan ou la mer, où elles vont contribuer à la pollution microplastique. Le complément

Nous espérons que, quatre années ayant passé, les consciences auront évolué et que cet amendement pourra être adopté. Les faits sont têtus : selon une étude de l'ONG 5 Gyres, environ 268 000 tonnes de plastiques flottent aujourd'hui dans les océans du globe,

de polytéréphtalate d'éthylène, de polyméthylméthacrylate ou de nylon. Les microbilles ne sont pas uniquement utilisées pour leurs vertus exfoliantes et nettoyantes, mais également pour en tant qu'agent de polissage, pour leurs effets émulsifiants comme volumificateurs, pour leurs propriétés filmogènes filmogènes ou pour réguler la viscosité des produits. Après utilisation, les microbilles de plastique s'écoulent par le drain de douche ou l'évier dans les réseaux d'eaux usées et les égouts. Elles sont trop petites pour être retenues par les par les filtres des stations d'épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d'eau, pour finir leur course dans l'océan ou la mer, où elles vont contribuer à la pollution microplastique. Le complément de rédaction que nous proposons permettrait d'élargir le champ des produits visés, en y incluant notamment

rectifié. Une fois de plus, je souhaite rappeler que la commission a adopté des dispositions permettant de faire financer par les producteurs de ces produits des opérations de nettoyage des milieux et de traitement de la pollution des eaux.

les objectifs ambitieux que nous avons fixés : 100 % de plastique recyclé en 2025, diminution de la mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique et réduction des déchets ménagers.

La production, le transport, la transformation et le recyclage de certaines matières plastiques de l'industrie pétrochimique, comme les granulés et paillettes de plastique, conduisent à des pertes de confinement. Ces déchets, répandus à l'échelle mondiale, échappent aux opérations régulières ou exceptionnelles de ramassage et constituent un risque avéré de contamination des chaînes alimentaires marines,

ces petits granulés sont partout présents. Il convient d'améliorer les conditions de confinement pendant la fabrication, la transformation et le transport multimodal. En 2016, 60 % des plages surveillées étaient polluées par les granulés de plastique industriels, la concentration pouvant atteindre 40 000 grains au mètre carré dans certains comme l'estuaire de la Seine. L'industrie prend des initiatives, telle l'opération Clean Sweep, mais, en l'absence d'un audit indépendant, il n'existe que peu d'informations sur leur efficacité. Il est nécessaire de renforcer les systèmes d'emballage, de stockage et de transport de ces granulés de plastique industriels, en optant pour des fûts rigides à ouverture totale avec fermeture hermétique, et d'y indiquer la mention « dangereux pour l'environnement ». Seul un étiquetage adéquat permettra la sensibilisation et la formation des gestionnaires des routes, des voies de chemin de fer et des services de secours et de sécurité publique à ces déversements accidentels de produits chimiques

Nous avons engagé un travail avec les représentants de la plasturgie pour que ceux-ci s'engagent à rendre compte des actions mises en oeuvre dans le cadre du programme Opération Clean Sweep, qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique. Nous devons dresser un premier bilan de ce programme afin d'identifier les mesures les plus pertinentes et de déterminer les actions les plus